Mes chers collègues, le projet de loi confortant le respect des principes de la République a été envoyé pour examen à la commission des lois. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication et la commission des finances ont demandé qu'il leur soit renvoyé pour avis.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

par le directeur sur proposition du président de la CME, sans que les postulants soient nécessairement membres de cette dernière. Le rôle du directoire est d'accompagner le directeur par la concertation dans la conduite de la politique de l'établissement. Le Gouvernement semble fonder les dispositions qu'il propose sur les réserves émises par le professeur Claris sur le directoire. Or celles-ci visent non pas l'utilité du directoire dans la gouvernance hospitalière- il est rappelé que c'est une « instance essentielle » -, mais les liens qui doivent être entretenus entre lui et les praticiens hospitaliers de terrain.

la possibilité pour le directeur de procéder à la nomination de « personnalités qualifiées » susceptibles d'être choisies hors du personnel de l'établissement sans autre critère de sélection. concerne la présence des étudiants, la conférence nationale des directeurs de centre hospitalier (CNDCH) a relevé que les étudiants exerçaient « très temporairement » dans les établissements et que leur apport réel sur la stratégie de l'établissement ne pouvait qu'« être limité, sachant qu'il est jugé mince au sein des CME

Poncet Monge. Le Ségur de la santé a souligné la nécessité de prendre en compte les différents acteurs de la santé et d'améliorer le dialogue au sein de l'hôpital. L'article 9 va dans ce sens, en permettant l'intégration des usagers et des étudiants en santé dans le directoire. Nous nous félicitons d'une telle avancée. En effet, le directoire appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement et de son projet. Il est logique que chaque acteur de la santé y prenne sa place, car aucune catégorie ne peut prétendre représenter à elle seule l'intérêt général. C'est précisément la pluralité des points de vue, des « lieux d'où l'on parle », qui permet de faire émerger des décisions pertinentes. Mais, en l'état actuel du texte, cette présence n'est qu'une possibilité laissée à la seule discrétion du directeur. Nous proposons d'intégrer la reconnaissance de l'intérêt de la présence des représentants des usagers et des étudiants, en la rendant systématique. Intégrer systématiquement les représentants des usagers dans le directoire permettra de mieux appréhender les besoins de la population, à qui s'adresse le service public de santé. Cela enverrait un signal fort de démocratie sanitaire. Intégrer systématiquement les étudiants en santé

Cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise donc à rendre obligatoire la présence des représentants des usagers et des étudiants en santé au sein du directoire, d'autant que leur voix- je le rappelle -reste consultative. Quel

que les agences régionales de santé doivent être une boîte à outils pour accompagner les hôpitaux. Or, dans la réalité, elles sont le bras armé de Bercy et de la réduction des dépenses, en imposant des fermetures de lits et la réorganisation des services.

de pénalités financières : les donneurs d'ordre ne peuvent pas être aussi les contrôleurs financiers. Nous proposons donc la suppression des pouvoirs de sanction financière des ARS. Quel est l'avis

En effet, le développement des compétences sanitaires des régions constitue une attente forte des élus locaux. Les régions interviennent dans l'organisation du parcours de soins à travers la définition du schéma régional de santé. Elles sont également compétentes en matière de

il apporte des précisions budgétaires sur deux points. D'abord, le montant journalier des dépenses susceptibles d'être engagées au titre du travail temporaire devra obligatoirement figurer à l'EPRD. Ensuite, le directeur général de l'ARS, s'il constate que ce montant dépasse le plafond défini par décret, renverra l'EPRD au directeur d'établissement et réservera son approbation jusqu'à ce que ce montant soit inférieur au plafond. À l'issue de l'exécution du budget de l'établissement, si le compte financier fait apparaître un dépassement du plafond, le directeur général de l'ARS devra déférer au tribunal administratif

Ces deux dysfonctionnements relevant de ses compétences, nous demandons simplement que le déontologue de l'hôpital soit également informé, au même titre que le directeur d'établissement et le conseil de surveillance. Cet ajout ne modifie en rien le process établi par le rapporteur, dont nous venons de discuter.

Le premier permet de liquider la dette de l'ordonnateur vis-à-vis d'un prestataire ayant déjà fourni un service, tandis que le second s'exerce en amont de l'engagement afin d'en vérifier la régularité.

lié au rôle que tout représentant de l'État dans un territoire doit exercer au regard de l'application de la loi. Cette déresponsabilisation n'a pas paru souhaitable à la commission des affaires sociales. Nous avons donc émis un avis défavorable sur l'amendement de rétablissement du Gouvernement, en souhaitant évidemment que nous puissions tous ensemble en rediscuter dans le cadre de la

part, je serais tentée de vous alerter en amont sur le fait que vous êtes en train de produire la même situation dans le monde médico-social.

il me semble que nous ne sommes pas en mesure, même sur les moyen et long termes, de remédier suffisamment à ce problème. Cette question, au-delà des hôpitaux et des déserts médicaux, devient tout à fait insupportable pour nos concitoyens et devrait malheureusement avoir

Cet amendement vise à rétablir l'article 11, en ajoutant un volet numérique dans le projet d'établissement afin de répondre aux besoins d'interopérabilité. Tout d'abord, le projet de gouvernance et de management semble un outil pertinent qui était recommandé par le rapport Claris. En effet, ce document permettra de définir les orientations stratégiques, notamment en matière de gestion des équipes médicales, paramédicales et administratives. Il assurera également la prise en compte des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l'accompagnement des étudiants en santé.

Afin de permettre que l'investissement dans le numérique puisse être utile au plus grand nombre et dans un objectif de simplification du système de santé, prendre en compte le numérique est central.

Or, pour cette année de transition et pour respecter le droit au redoublement dans l'ancien système Paces, des places sont réservées aux redoublants au regard de la capacité totale par faculté, ce qui rend le taux de réussite pour les étudiants en PASS proche de 10 %. Voilà qui va totalement à l'inverse

dans la plupart des facultés, sans augmentation du nombre de places et avec de surcroît un programme très lourd et une licence à valider. En outre, si, pour les redoublants de la Paces, la seule contrainte pour redoubler était de s'inscrire, il n'en est rien pour les étudiants en PASS

Ils ont dénoncé des comportements sexistes, racistes et homophobes à l'hôpital. Ainsi, 93 % des étudiantes en médecine générale déclarent avoir subi des violences psychologiques, 53 % des violences sexuelles et sexistes,

qui jette l'opprobre sur l'ensemble des personnels hospitaliers, ce qui est profondément injuste. Nous avons rencontré des responsables de l'Association nationale des étudiants en médecine de France

partagé par l'ensemble de l'hôpital. C'est le sens de cet amendement qui vise à inscrire directement la lutte contre le racisme, le sexisme et l'homophobie dans les objectifs du projet social de l'établissement. Actuellement, ce projet social définit des objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement, ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, le dialogue interne au sein des pôles, le droit d'expression des personnels et sa prise en compte,

de psychologues coordonnateurs pour clarifier son organisation et son fonctionnement.

Historiquement autorisée pour apporter un complément de rémunération aux médecins, notamment en prévision de leur retraite, cette activité privée augmente pour une minorité de médecins concernés. Une enquête du magazine a montré une tendance en progression au fil des années. Ainsi, en 2016, 2 181 médecins hospitaliers ont facturé 70 millions d'euros de dépassements d'honoraires dans le cadre de leur activité privée à l'hôpital sur les 4 722 médecins hospitaliers autorisés à exercer une activité privée à l'hôpital public, près de la moitié sont installés en secteur 2. Je rappelle que nous ne sommes pas du tout opposés à cet exercice mixte,

34 000 infirmiers et 24 000 aides-soignants. Cette augmentation doit s'appuyer sur les besoins définis en région, notamment dans le cadre du schéma régional des formations sanitaires. Il est proposé que ce schéma s'appuie sur l'évaluation des besoins

On peut d'ailleurs saluer l'intérêt pour ces structures des articles 12 et 13 du texte. Toutefois, je souhaiterais apporter une précision technique. Les améliorations pérennes sur les modalités de gouvernance proposées par l'article 13 pour les mutuelles du code de la mutualité doivent avoir leur pendant dans le code des assurances. De ce fait, il semble logique, cette fois par voie réglementaire, que les dispositions de l'article 13 trouvent un prolongement pour les mutuelles d'assurance. En effet, si les mutuelles sont régies par des règles issues de deux législations distinctes, elles partagent les mêmes modes d'organisation. Telle est l'information que je souhaitais vous apporter, monsieur le ministre.

L'article 14 prévoit la création d'une plateforme numérique nationale d'information et de services personnalisés destinée aux personnes en situation de handicap. C'est une réelle avancée. Il conviendra toutefois de bien veiller à ce que sa mise en oeuvre ne se fasse pas au détriment de l'accueil physique et téléphonique, comme cela est d'ailleurs précisé dans le texte. Plusieurs amendements sont venus enrichir cet article pour garantir l'accessibilité de cette plateforme. Nous nous en félicitons également. La Caisse des dépôts et consignations se verra confier la gestion de la plateforme. Il est précisé qu'elle devra collecter le retour d'expérience des utilisateurs pour améliorer en continu son utilisation. Cette mention est bienvenue, mais elle est insuffisamment inclusive. Cette plateforme, qui a pour vocation de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap, de leurs aidants et de leurs représentants légaux doit être construite

C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose, par cet amendement, que la création et la gestion de la plateforme s'effectuent en collaboration continue avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), afin de prendre en compte au mieux les préoccupations et les problématiques des usagers et de leurs représentants.

». S'il s'agit d'associer le CNCPH à la conception des services proposés sur la plateforme, l'amendement est satisfait, car il fait partie du comité des parties prenantes installé formellement par Mme Cluzel le 10 décembre 2020.

au service numérique de la plateforme est assuré par le département.

n° 12 rectifié. Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes soins que l'ensemble de la population. Le handicap ne peut être un critère de refus de soins, qu'il s'agisse d'hospitalisation ou de réanimation. L'axe « handicap » du Ségur de la santé a pointé la nécessité de lancer un programme d'adaptation des conditions de soins pour les personnes handicapées. La Haute Autorité de santé (HAS), dans son guide « Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap », met en exergue comme bonne pratique

au collectif Handicaps. Par cette précision législative, les représentants des usagères et des usagers porteurs de handicaps entendent faire valoir leur droit à la différence dans les soins qui sont dispensés à l'hôpital. Ces personnes nous disent en effet qu'elles ont des besoins particuliers

recommandait en effet de mettre en place un référent « handicap » afin d'accueillir les patients, quel que soit leur handicap, et de les accompagner à chaque étape de leur parcours de soins. C'est d'ailleurs une idée qui a fait son chemin dans le monde de l'entreprise, puisque, sur l'initiative du député Adrien Taquet, son avenir professionnel de septembre 2018 a rendu obligatoires de tels référents « handicap » dans les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés. Reste à préciser le maillage opportun. Le guide de la HAS préconisait un référent par établissement

et les besoins d'accès aux soins de la population, alors que l'ensemble des spécialités médicales est financé par la solidarité nationale. Il a également vocation à rattraper les inégalités de traitement

pour déplorer que ce texte, qui était jugé, de manière quasi unanime, peu ambitieux, ait été amputé de mesures qui nous semblaient intéressantes. Je pense évidemment aux auxiliaires

Pour autant, il serait malhonnête de rejeter en bloc le travail du Sénat, de la commission des affaires sociales et, bien sûr, de notre collègue rapporteur. Il serait dommage également de s'opposer à un texte, même modifié, qui va globalement dans le bon sens. C'est pourquoi le groupe RDPI s'abstiendra, à regret, sur cette proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. La parole est à M.

ce texte. Sur le reste, nous n'avons pas vraiment pu échanger avec le Gouvernement et je le regrette. Ce texte reste marqué des défauts que nous pointions dans la discussion générale,

pour nous donner quelques semaines de plus, le temps de prendre connaissance de l'ordonnance qui sera publiée sur la question au mois de mars. Nous aurions alors pu légiférer avec une meilleure visibilité. Ensuite, nous restons sur l'idée que cette proposition de loi a toutes les caractéristiques d'un projet de loi et qu'un avis du Conseil d'État aurait été nécessaire. Les discussions que nous avons eues ont parfois montré une difficulté à appréhender

de notre système de santé, c'est avant tout en tirant les leçons de l'épidémie qui nous frappe et qui a mis en lumière les défauts de notre système de santé public. Or on ne trouve aucune réponse dans ce texte. Est-ce trop tôt ? Non ! Il est temps,

vote. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur la nature de ce texte.

et l'ensemble des soignants, qui attendent vraiment qu'on fasse bouger les choses. Merci encore une fois pour l'ambiance dans laquelle ce travail s'est déroulé ; je suis vraiment ravi d'avoir pu y participer autant que possible.